La séance est reprise. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres,

Cette année encore, un conglomérat chinois a confirmé à la mi-février avoir racheté environ 3 000 hectares pour cultiver du blé. Les fariniers chinois semblent très sensibles à la réputation du blé français. Nous pourrions nous en réjouir, mais cette pratique pose problème à plus d'un titre. Tout d'abord, les fonds de gestion chinois transforment l'exploitation en société, pour contourner le contrôle opéré par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les SAFER. Par ailleurs, ces rachats de terres se font auprès d'exploitants endettés, à des prix trop élevés pour que de jeunes agriculteurs puissent reprendre ces terres. Enfin, une fois nos terres cédées, la production est destinée à l'exportation. Depuis 2016, le législateur a tenté de remédier à ces pratiques en élargissant le contrôle des SAFER sur la cession des parts, mais uniquement si 100 % des parts sont mises en vente. Le contournement est facile : les cessions de parts se font à hauteur de 98 D'autres tentatives d'évolution de notre législation par le Parlement n'ont pas abouti. Pour autant, nous ne devons pas nous résigner. L'enjeu est trop important et peut, à terme, se révéler crucial pour notre souveraineté Monsieur le ministre d'État, le Président de la République a annoncé la mise en place de « verrous réglementaires » sur les achats de terres agricoles par des étrangers. Qu'en est-il ? Comment comptez-vous faire pour protéger notre indépendance

l'achat récent de terres agricoles françaises par des sociétés étrangères suscite un grand émoi et de nombreuses interrogations- nous en avons, bien évidemment, tout à fait conscience. Toutefois, avant d'évoquer un phénomène d'accaparement des terres, il faut examiner la réalité des données.

difficile, à ce stade, de parler d'un phénomène d'accaparement des terres ; ces opérations relèvent plus de stratégies d'investissement, comme peuvent le faire nos opérateurs à l'étranger. Néanmoins la vigilance et la transparence doivent être de mise- c'est en ce sens que le Gouvernement

paraissent clairement inadaptés face au développement d'opérations conduites sous forme sociétaire et pouvant aboutir à des phénomènes de concentration. Les récentes évolutions législatives ont permis d'améliorer le dispositif, avec un droit de préemption accordé aux SAFER pour l'acquisition de la totalité des parts sociales d'une société dont l'objet principal est la propriété agricole. Mais nous constatons

Au cours du précédent quinquennat, plusieurs mesures n'ont fait que complexifier un système assurantiel déjà illisible pour nos concitoyens et affaiblir les droits de ces derniers pour leur couverture santé. Je pense à la loi du qui a généralisé les réseaux de soins. Dans ce cadre, possibilité a été donnée aux complémentaires dans les trois secteurs- optique, dentaire, audioprothèse -de différencier les remboursements en fonction du choix de son professionnel. Nous l'avions dénoncé. Je pense également à l'obligation des contrats collectifs pour tous les salariés, qui a dégradé la couverture assurantielle des contrats individuels des inactifs, notamment des retraités, et qui s'est traduite par une pression fiscale supplémentaire de près de 1 milliard d'euros par an pour les salariés, avec la fiscalisation de la part employeur. Enfin, le plafonnement du remboursement des soins médicaux des contrats responsables obtient la palme, puisque c'est le contrat qui rembourse le plus mal et qui est deux fois moins taxé par l'État. Une étude, fort enrichissante, de l'UFC-Que choisir fait ressortir le coût toujours plus important des complémentaires de santé dans le budget des Français. Ce coût a progressé trois fois plus vite que l'inflation au cours de la dernière décennie. En 2016, la Cour des comptes avait, d'ores et déjà, déploré des dépenses de 7,2 milliards d'euros en frais de gestion, dont près de 3 milliards d'euros pour la publicité. La réforme sur le reste à charge zéro et la remise à plat du secteur des complémentaires de santé, madame la ministre, ne sont que les deux facettes d'une même médaille : vouloir les traiter séparément, c'est prendre le risque de faire peser de plus en plus la part des cotisations des assurances de santé sur le budget des ménages. C'est pourquoi je souhaite connaître les mesures que vous pensez adopter pour encadrer la lisibilité des offres des complémentaires de santé et exiger une meilleure transparence sur les frais de gestion.

vous le savez, les complémentaires de santé sont essentielles pour l'accès aux soins des Français : 95 % de nos concitoyens sont couverts, soit par une complémentaire de santé, soit par la

en fonction du soin remboursé. Notre objectif est bien que la réforme n'induise aucune augmentation de tarif. C'est un point ayant fait l'objet de nombreux échanges avec les fédérations d'organismes complémentaires, et sur lequel nous serons particulièrement vigilants. Nous avons prévu un comité de suivi de la réforme, qui se

de placer les recettes de ces ventes dans un fonds, dont le rendement servirait à financer l'innovation des entreprises. Si nous souscrivons à l'objectif, la méthode interroge. Nous avons ici des entreprises rentables, qui prospèrent et versent chaque année jusqu'à 1 milliard d'euros de dividendes, contribuant ainsi au financement de l'État et de la dette. Des entreprises qui exercent dans des domaines stratégiques en forte croissance, pour lesquels un pilotage étatique se justifie- transport aérien, régulation des jeux ou encore transition énergétique. l'heure où l'État doit non pas seulement diminuer ses dépenses, mais aussi consolider ses recettes, quel intérêt y a-t-il à vendre des actifs rentables et renoncer à des rentrées d'argent récurrentes ? D'autant que ce fonds stratégique- important -pourrait être financé d'une autre manière, par emprunt, les dividendes annuels évoqués permettant de financer les annuités. En définitive, ce fonds serait disponible, les entreprises innoveraient et les Français seraient toujours les heureux propriétaires d'ADP, FDJ et Engie

Monsieur le secrétaire d'État, à force de nationaliser les déficits et de privatiser les bénéfices, nous appauvrissons l'État. Vous avez parlé d'innovation pour l'avenir. L'innovation, notamment dans l'administration de la France, c'est peut-être aussi inventer de nouveaux partenariats gagnants-gagnants,

Nous approchons de la période où vont se clore les discussions, avec 322 grandes collectivités territoriales, sur les contrats permettant de maîtriser, d'un commun accord, l'évolution des dépenses de fonctionnement.

Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous indiquer quel est l'état des conclusions d'accords envisagées par les collectivités et les points restant en discussion avec certaines d'entre elles ? Je pense, en particulier, au sujet spécifique des collectivités connaissant une forte croissance démographique, mais aussi à certaines catégories de dépenses qui sont exposées par les collectivités, sur la suggestion de l'État et, d'ailleurs, avec son aide.

entre les 322 principales collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale et l'État -, nous essayons d'inventer d'inventer une nouvelle façon de travailler et de maîtriser l'augmentation de la dépense publique locale, c'est-à-dire un nouveau mode de fonctionnement entre les collectivités territoriales et l'État. Chacun se souvient ici qu'il fut un temps, pas si lointain, où les contraintes générales

L'idée est d'encadrer l'augmentation de leurs dépenses de fonctionnement, à un taux moyen de 1,2 %. C'est un exercice nouveau et, évidemment, il est particulier

Nous avons entendu ces remarques. Nous avons créé des critères de modulation en fonction de l'évolution de la population et d'un certain nombre d'indicateurs. Nous avons également indiqué, aux collectivités qui le souhaitaient, que

aux demandes formulées par les régions, parce que nous considérions que, ce faisant, nous restions dans l'épure, dans le sens même de cette contractualisation qui avait été engagée.

une véritable crise européenne s'est ouverte sur le sujet, à la suite de plusieurs évènements récents. D'une part, le refus total du nouveau gouvernement italien d'accueillir les 629 migrants de. D'autre D'autre part, l'ultimatum posé par le ministre de l'intérieur allemand, Horst Seehofer, à la chancelière Angela Merkel, lui intimant de réduire substantiellement le nombre de migrants accueillis en Allemagne, sous peine de refouler aux frontières ces mêmes migrants. Cette crise politique interne pourrait avoir des conséquences importantes sur la politique migratoire européenne. Nous savons, monsieur le ministre d'État, que vous avez participé avec le Président de la République à un conseil des ministres franco-allemand, ce mardi, pour trouver un consensus et arrêter une position commune. De même, sur invitation du président Jean-Claude Juncker, M. Emmanuel Macron participera, ce dimanche, à une réunion de travail, certes informelle, sur le sujet, pour débloquer la situation en amont du Conseil européen des 28 et 29 juin. Ce conseil s'annonce déjà difficile, la Commission européenne proposant de réformer le règlement de Dublin, en instaurant notamment une répartition automatique des demandeurs d'asile dans l'Union européenne en période de crise comparable à celle de 2015. Monsieur le ministre nous le savons tous, les réponses apportées à la question migratoire ne peuvent qu'être européennes. Dans ce contexte tendu, pouvez-vous éclairer la représentation nationale sur la situation politique en Allemagne et sur l'avenir de la politique migratoire européenne ? Pouvez-vous nous assurer que la France fera tout pour parvenir à un accord acceptable et respecté par tous les États membres ? Sinon, il est à craindre un affaiblissement de l'Union européenne, que nous avons mis tant de temps à construire.

citerai d'abord l'accord conclu entre l'Union européenne et la Turquie, qui a évidemment fait baisser de manière considérable

Et c'est la première fois depuis un an et demi que l'on voit de nouveau des bateaux chargés de migrants ! Oui, vous avez raison, la solution sera européenne. Nous allons y travailler. Le Président de la République y oeuvrera dimanche prochain, afin de trouver un accord européen

Pour amplifier la contribution des collectivités locales à la réduction des déficits publics, le Président de la République et le Gouvernement ont clairement changé de méthode, mais pour atteindre le même objectif 13 milliards d'euros que s'élève le montant de la nouvelle réduction des dépenses utiles que vous avez décidé d'imposer aux services publics locaux d'ici à 2022, après les 11 milliards d'euros de baisse de dotations du précédent quinquennat. Vous avez mis en place un outil redoutable, au nom pour le moins abusif : les contrats État-collectivités. Oui, ce nom est abusif, parce que ces contrats sont construits sur des principes décidés par une seule des parties, à savoir l'État, et n'engageant en vérité que l'autre, les collectivités territoriales.

pour les collectivités qui ne se plieraient pas au 1,2 % d'évolution des dépenses de fonctionnement. Et, à ce titre, il est contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités.

quels sont précisément les bénéfices attendus de ces contrats imposés aux collectivités, pour les populations et pour les territoires ?

monsieur le sénateur Pascal Savoldelli, entre ce qui s'est passé les dernières années et ce qui se passe aujourd'hui, permettez permettez à l'ancien gestionnaire de collectivités locales

de 8 % en 2014, de 8 % en 2015, du fonctionnement de 0,2

nous avons fait les calculs pour les différentes strates de collectivités, et c'est pour cela que 60 % des collectivités vont signer le pacte que nous leur proposons.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Mme la ministre des solidarités et de la santé. À l'heure où le Président de la République s'insurge contre le « pognon de dingue » versé à nos concitoyens les plus modestes et en appelle à « la responsabilisation des pauvres », je souhaiterais vous interroger sur ce sujet, car il est grave et mérite mieux que des formules aussi scandaleuses que dangereuses pour notre contrat social. Cette musique droitière, nous la connaissons. Vous cherchez à démontrer que les minima sociaux ne « fonctionnent pas » en vue de préparer les coupes budgétaires à venir, évaluées à 7 milliards d'euros par Bercy : c'est le montant des cadeaux fiscaux aux plus fortunés. D'autres acteurs, plus responsables, en prise avec les réalités de notre pays, imaginent les solidarités de demain. Je pense notamment aux treize départements socialistes qui ont mis sur pied un projet d'expérimentation d'un revenu de base. Leur proposition est simple : offrir aux citoyens vivant sous le seuil de pauvreté une allocation qui fusionnerait le RSA, la prime d'activité et potentiellement les aides au logement. Ce projet présente l'avantage de traiter la question majeure du non-recours aux aides sociales, de simplifier le système de prestations et de lutter efficacement contre la précarité. Bien sûr, ce programme d'éradication de la grande pauvreté ne pourra se faire sans argent public pour être expérimenté à grande échelle. Madame la ministre, êtes-vous prête à soutenir cette initiative originale lors de l'examen des projets de loi de finances ? Vous semblez déjà évoluer vers un renforcement de l'expérimentation « territoires zéro chômeur » lancée sous le précédent quinquennat. En sera-t-il de même pour cette nouvelle expérimentation ambitieuse ? Avez-vous pris la mesure de « l'urgence à agir » en matière de lutte contre la pauvreté ?

le RSA -et de porter une attention particulière à la pauvreté des jeunes. Cependant, ces expérimentations ne posent pas les bonnes questions. Leur objectif notamment nous interroge : voulons-nous attribuer à chaque personne en situation de pauvreté une allocation monétaire pour solde de tout compte ? Le projet du Gouvernement est totalement différent : il est global pour mieux prendre en compte la situation réelle des personnes. Nous voulons travailler sur la question des freins périphériques au retour vers l'emploi et renforcer le rôle incitatif des prestations. Aujourd'hui, nous le savons, nos aides sociales sont inéquitables, différentes selon le statut et selon l'âge, illisibles- c'est un maquis, aucun d'entre nous, aujourd'hui, ne sait les citer -, insuffisamment tournées vers l'accompagnement. Notre souci, c'est de prévenir la pauvreté à toutes les étapes de la vie, de l'enseignement primaire- c'est ce que fait Jean-Michel Blanquer avec le dédoublement des classes de CP, le plan Mercredi, le plan Devoirs faits -jusqu'à l'insertion sur le marché du travail, à laquelle Muriel Pénicaud travaille avec avec la réforme de la formation professionnelle. La première arme de lutte contre la pauvreté, c'est l'accès à un diplôme, à une qualification. Nous voulons mettre un terme au déterminisme social, aux situations qui enferment les personnes dans l'inactivité ou la sous-activité. Nous ne voulons plus nous contenter d'une politique d'insertion qui ne permet qu'à 10 % des allocataires du RSA de retrouver une activité chaque année. Notre projet, c'est bien l'efficacité et l'investissement humain, dans lequel nous misons toutes les forces de la Nation. La parole Madame la ministre, sans les transferts sociaux et fiscaux, notre pays compterait 5 millions de pauvres supplémentaires. La redistribution est au coeur de notre fraternité et fait la force de notre modèle social. Après un an d'exercice du pouvoir, le résultat de votre politique s'avère foncièrement injuste. Vous parlez d'émancipation sociale, mais, en catimini, vous baissez une nouvelle fois les APL pour les plus pauvres. Vous vantez les modèles allemand et britannique alors que leur taux de pauvreté est bien supérieur au nôtre. Le revenu de base est un bon outil pour lutter contre l'exclusion sociale, saisissez-le

Cette question est un cri d'alarme. En 2010, la loi sur le Grand Paris a défini un objectif très ambitieux de production de 70 000 logements par an en Île-de-France. Pour atteindre cet objectif, le triptyque logement-développement était le fondement du contrat de confiance liant l'État et les collectivités territoriales. En confiance donc, les collectivités ont rempli leur part du contrat. Le département des Yvelines, que vous connaissez bien a ainsi produit de façon volontariste 12 000 logements par an depuis dix ans. Oui, nos maires sont tous des bâtisseurs ! De son côté, l'État s'était engagé à construire des infrastructures de mobilité : des routes, des parkings de rabattement, le Grand Paris Express, la ligne pour la partie ouest. Où sont les promesses de l'État ? Les infrastructures de mobilité sont tellement saturées qu'un léger dysfonctionnement fait basculer en enfer la matinée de millions de travailleurs pendulaires. La semaine dernière est emblématique : A 13 fermée car inondée ; gare Saint-Lazare en total black-outRER A en panne ; RER B déraillé ; grèves de la SNCF ... Mais cette situation est en réalité notre quotidien : un simple accrochage sur l'autoroute ou un incident voyageur débouche sur une thrombose généralisée. Pourtant, nous devons continuer à construire, sans faiblir, sans solution de mobilité. Alors, monsieur le Premier ministre, je ne vous rends naturellement pas coupable ou responsable de ce chaos. Mais vous incarnez l'État et êtes aujourd'hui comptable de ses engagements. Vous avez pris la décision de retarder la réalisation de grandes infrastructures de mobilité, alors allez jusqu'au bout et revoyez avec les élus le calendrier de leurs obligations à construire. Je vous le demande sans esprit de polémique mais fermement, car ajouter la thrombose à la thrombose conduit à l'incompréhension, à la désespérance et peut-être à la révolte de nos concitoyens

s'est donné les moyens à la fois financiers et opérationnels de rendre possible ce futur métro. Ils y croient ! La confiance entre l'État et les collectivités, c'est se donner un calendrier qui soit réaliste et tenir les promesses, mais les tenir avec sincérité. Le Premier ministre a confirmé l'intégralité du tracé du Grand Paris Express

Le Gouvernement souhaite également s'assurer du financement de ce projet majeur. À ce titre, il a confié une mission au député Carrez pour stabiliser les recettes de la Société du Grand Paris, maître d'ouvrage des opérations. ! Enfin, notre gouvernement a aussi pris le parti du réalisme en tenant compte des retards inéluctables dans le cours des opérations de construction. Ce réalisme participe de la confiance entre les parties. Vous évoquez également la question du logement. Le Grand Paris Express est un acteur majeur de la transformation urbaine : il doit participer à la mutation des quartiers et à la production des logements en Île-de-France. Ainsi, ce sont 600 000 mètres carrés de bâti qui sont prévus ou à l'étude autour des gares. Mais, pour autant, à date, seuls huit projets immobiliers liés directement aux gares étaient déjà attribués. De nombreux autres projets sont à l'étude et seront installés autour des infrastructures que nous bâtissons. Comme je vous le disais en introduction, madame la sénatrice, le recalage du calendrier n'implique aucun abandon de desserte de métro. De la même manière, les projets de logements accompagneront ce nouveau calendrier. pour la réplique. Madame la Première ministre, je vous remercie de cette réponse, qui montre le mépris que vous avez pour les élus locaux. Vous répondez totalement à côté de la question La parole est à Mme Lana Tetuanui, pour le groupe Union Centriste. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, '! Monsieur le Premier ministre, consultée le 7 juin, l'Assemblée de Polynésie française a émis à l'unanimité des courants des courants politiques un avis défavorable sur le futur volet organique et ordinaire de la réforme des institutions. D'une part, la réduction du nombre de parlementaires a été jugée inefficiente en Polynésie du fait de notre configuration géographique

Il s'agit, à mon sens, et je pèse mes mots, d'une régression, voire d'un muselage démocratique. Et que dire de nos frères Et que dire de nos frères calédoniens ? Votre projet de réforme passe mal, car nos collectivités présentent des particularités qui n'existent ni en France métropolitaine ni dans les DOM, et parce que le droit permet une adaptation des dispositions législatives et réglementaires pour prendre en compte nos spécificités. Étant donné leur situation géographique, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ne peuvent se réduire uniquement à des considérations d'ordre démographique Je tiens à rappeler les enjeux géopolitiques stratégiques de la zone Pacifique, que le Président de la République a bien voulu signifier lors de son dernier passage en Australie et en Nouvelle-Calédonie, qualifiant la France de grande puissance de l'Indo-Pacifique à travers ses collectivités ultramarines, où la représentation nationale doit être privilégiée et consolidée dans l'intérêt de notre nation. pourriez-vous me rassurer sur la prise en compte de nos spécificités géographiques, afin de représenter au mieux les intérêts de la République française dans notre région du Pacifique ? La parole

la prise en compte des particularités de chaque territoire d'outre-mer est une priorité du Gouvernement. C'est le sens du droit à la différenciation voulue par le Président de la République, c'est le sens de la révision de l'article 73 de la Constitution proposée par le Gouvernement, c'est le sens de l'accompagnement des évolutions statutaires souhaitées par plusieurs territoires et par le ministère des outre-mer, et la Polynésie française est concernée. est concernée. Tous ces éléments seront rappelés dans le livre bleu des outre-mer, qui sera rendu public jeudi. Mais certains principes, certains engagements politiques ne peuvent faire l'objet de dérogations territoriales, parce que cela aboutirait tout simplement à les remettre en cause.

jours, par exemple en confirmant l'engagement fort du Gouvernement pour la santé des Polynésiennes et des Polynésiens. Il l'a aussi rappelé en évoquant un signe fort qui vient d'être donné en faveur du développement du numérique, qui est une réponse particulièrement adaptée à l'étendue de votre territoire. Nous nous attachons, et vous le savez, avec le Pays, avec les parlementaires, à entretenir un dialogue de confiance, un dialogue constant. Blablabla ... Mais l'engagement du Président de la République pour une démocratie représentative, efficace et responsable concerne l'ensemble des parlementaires, dont le nombre diminuera dans chaque assemblée de 30 %. S'il est mis en oeuvre partout, le projet de loi contient des garanties permettant une représentation juste des territoires. D'ailleurs, il sera bien sûr contrôlé par le juge constitutionnel. Ainsi, le projet de loi

En outre, les critères de redécoupage de 2009 sont repris et même renforcés. Il faut conclure. Madame la sénatrice, parce que les Français en ont exprimé la volonté, une modernisation de nos institutions et de nos pratiques politiques sera faite sur tout le territoire.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de l'action et des comptes publics. Monsieur le ministre, le 1 mai dernier, le Président de la République a annoncé la suppression prochaine de l'. Celle-ci cible depuis 2012 les contribuables qui seraient tentés de s'exiler fiscalement afin de vendre leur société ou leurs participations sans s'acquitter d'un impôt sur la plus-value. Les personnes détenant au moins 50 % d'une société ou 800 000 euros de titres et se domiciliant fiscalement hors de France sont visées. Quinze années après leur départ, elles ne seront plus assujetties à la taxe. Avant cette échéance, la valeur prise par leur patrimoine entre son acquisition et leur départ de l'Hexagone fera l'objet d'une imposition en cas de cession. Le Président de la République, pour justifier son choix, a notamment mis en avant le faible rendement de l'impôt. Mais l'est Mais l'est un impôt dissuasif. Et si son rendement est faible, c'est justement parce qu'il remplit son objectif ! Le coût « véritable » de l'extinction de cette taxe- le manque à gagner pour l'État en cas de cession à l'étranger -serait de 2,5 milliards d'euros selon le Gouvernement. Ce chiffre a été revu fortement à la hausse la semaine passée par le responsable de la direction de la législation fiscale, qui l'estime désormais à 6 milliards d'euros. Monsieur le ministre, la suppression de l'ne nous paraît de l'ne nous paraît pas souhaitable. Il s'agit de l'une des rares barrières mise en oeuvre pour limiter l'optimisation fiscale. Sa suppression pourrait engendrer un appel d'air de départs à l'étranger pour vente de titres, dont les conséquences pourraient être beaucoup plus coûteuses pour l'État que les chiffres évoqués précédemment. Le chef de l'État a déclaré qu'il était pour l'idée de pouvoir se marier et d'être libre de divorcer ». Mais, monsieur le ministre, un entrepreneur doit aussi juger la réussite de son entreprise à l'aune de l'environnement économique et social que lui offre son pays. Nos compatriotes ne sauraient concevoir que le profit qui découle en partie de cet environnement puisse échapper ainsi à la solidarité nationale. Monsieur le ministre, comptez-vous toujours supprimer l'à compter de l'année prochaine ?

Jouve, l', c'est le génie français pour créer de la fiscalité, pour créer des barrières dont on oublie quelquefois que, parce qu'elles sont ouvertes, elles ne fonctionnent pas. L'consiste à faire payer à un entrepreneur qui s'installe à l'étranger un impôt sur les plus-values qu'il pourrait faire, si jamais il vendait les parts de son entreprise une fois expatrié.

dans l'industrie, 59 implantations de nouveaux sièges sociaux en France et 53 % d'augmentation des implantations de centres de recherche & développement. Madame la sénatrice, et je sais que c'est aussi le sens de votre question et de votre démarche, la France et tout faire pour renforcer son attractivité, c'est conforter nos emplois, nos économies, nos prélèvements sociaux et nos prélèvements fiscaux pour conforter nos caisses ! La parole

Je le dis d'emblée : je n'ai pas, et le groupe auquel j'appartiens non plus, d'opposition dogmatique à la privatisation. Je m'interroge davantage sur les arguments que vous avancez pour justifier ces cessions d'actifs. Par rapport à cela, j'ai trois interrogations. La première porte sur l'efficacité du privé par rapport au public. Les expériences en matière de privatisation des autoroutes me laissent sceptique sur ce point. En Allemagne, pays qui nous sert souvent de référence, le plus grand aéroport, celui de Francfort, est majoritairement détenu par la région et la ville. Est-il moins efficace ? Je ne le pense pas. La deuxième interrogation concerne le renforcement du rôle de l'État régulateur. Il paraît incongru de vouloir renforcer la régulation de l'État dans une entreprise en vendant ses parts. Vous évoquez le maintien de garanties. Mais quelle meilleure garantie que d'être actionnaire majoritaire ? Enfin, la troisième interrogation est relative au financement de l'innovation. À cet égard, nous sommes

moins que les dividendes actuels des entreprises visées ne rapportent à l'État ? Ma question est simple : quels sont les objectifs réels de ces privatisations ?

j'ai eu l'occasion de répondre partiellement dans la question précédente à vos différentes interrogations. Un bon actionnaire est un actionnaire qui sait se départir de ses habitudes. Une habitude pour un actionnaire est toujours une bien mauvaise chose. Croyez-moi, l'État, parfois par habitude, parfois par paresse, parfois par fainéantise, n'a jamais réinterrogé son actionnariat. L'objectif est donc, par ce projet de loi PACTE, de s'interroger sur les secteurs stratégiques et le rôle de l'État. Je réponds en cela à vos interrogations légitimes il n'est pas forcément utile d'être actionnaire d'une entreprise pour la réguler. Sinon, un grand nombre de secteurs dans lesquels l'État n'est pas actionnaire seraient mal régulés ; or, ce n'est pas le cas. On peut réguler sans être actionnaire, et on peut aussi renforcer les organismes de régulation sans être forcément actionnaire.

par Bpifrance de start-up. J'en ai assez de voir que figurent au fronton du CAC 40 français les mêmes entreprises depuis quarante ou cinquante ans quand, dans d'autres pays- je pense en particulier aux États-Unis -, l'essentiel des entreprises, et les plus grandes d'entre elles, n'existaient pas il y a quinze ans. Il est sain pour une économie

des choses qui vous ont rapporté 712 millions en 2017 ! Je me demande si l'objectif n'est pas plus simple : quand un gouvernement diminue les recettes de l'État et augmente les dépenses par des promesses non budgétisées,

Ma question s'adresse à Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé. Madame la ministre, le Président de la République a précisé dans son discours tenu devant les membres de la Mutualité sa vision de la société en termes de solidarité nationale. revanche, il n'a pas explicité sa politique familiale. Pourtant, la famille est au coeur d'une réforme sociétale qui se prépare : la réforme des retraites, dont je dois être le rapporteur.

Une question transgénérationnelle n'est pas précisée, celle de la pension de réversion, qui a été remise en cause dans certains pays, telle la Suède. Madame la ministre, ma question porte sur les pensions de réversion, symbole de la solidarité familiale affichée dans le régime actuel par répartition à prestations définies, mais qui pourraient être remises en cause dans une réforme future, par un régime par points, donc à cotisations définies, plus contributif que redistributif.

et de la santé. Mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Savary, le dispositif de réversion dont vous venez d'évoquer l'enjeu est un sujet de débat,

Vous le savez, il existe aujourd'hui 42 régimes de retraite différents, chacun ayant ses propres règles. Ces différences s'appliquent notamment aux pensions de réversion, dont les paramètres ne sont pas du tout les mêmes selon les régimes. Il est donc nécessaire de remettre à plat cette diversité de règles qui conduit aujourd'hui à de grandes injustices entre les Français, lesquels auront droit à des pensions différentes alors qu'ils sont confrontés au même drame, le décès de leur conjoint. À ces injustices s'ajoute une complexité importante : lorsque le conjoint décédé a été affilié à plusieurs régimes de retraite, chaque régime à son propre calcul et ses propres critères d'attribution, et le conjoint survivant doit engager des démarches souvent très longues et compliquées. Le résultat, en termes de montant perçu, peut varier considérablement d'un régime à l'autre. L'objectif de la concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux, telle qu'elle est menée par Jean-Paul Delevoye, est donc de refonder notre système de retraite en étudiant chaque dispositif, pas pour les supprimer, mais pour les harmoniser. Je terminerai en insistant sur deux points. La future réforme ne touchera pas les pensions déjà liquidées, bien entendu, et les personnes qui reçoivent déjà une pension de réversion ne verront aucun changement. Il n'est pas du tout non plus question de supprimer les pensions de réversion. Il s'agit simplement de repenser un dispositif pour qu'il soit plus juste, plus universel. La part de la solidarité restera la même dans la future réforme. La parole

une marque de la politique familiale, sur laquelle on juge un gouvernement. Cette politique familiale est trop souvent mise à mal et considérée comme une variable d'ajustement budgétaire ou fiscale. Pourtant, c'est bien le renouvellement des générations qui permettra de trouver un équilibre pour la réforme des retraites. N'oublions pas l'avertissement du général de Gaulle : sans le renouvellement des générations, la France ne serait plus « qu'une grande lumière qui s'éteint La parole est à M. Michel Vaspart, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. L'année 2017 aura vu une hausse de notre PIB de 2,3 %. C'est, pour la France, la plus forte croissance depuis 2007. Toutefois, ce taux, qui semble magnifique pour une économie qui n'a pas dépassé 2 % par an depuis dix ans, fait pâle figure au regard de la situation dans Monsieur le ministre, la France est à la traîne ! Sa croissance est médiocre et entravée par de multiples liens, impôts, taxes, surtranspositions de directives européennes, normes et excès de règlements, par l'incapacité de l'État à se réformer en profondeur réorganisation des collectivités locales, qui n'engendrent nullement des économies, mais entraînent des hausses, sans forcément apporter de services supplémentaires. Pour 2018, vous avez basé votre budget sur une croissance du PIB de 2 %. L'INSEE vient de baisser à 1,7 % la prévision de croissance. La consommation des ménages est faible, voire atone, le prix du pétrole remonte fortement, le contexte international se tend et nous attendons encore les réformes de fond. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour créer enfin dans notre pays un véritable choc de compétitivité de la France et en faire un véritable moteur, au service de nos concitoyens ?

nos politiques, nous partons tout simplement du constat. Nous l'avons fait sur le droit du travail, nous le poursuivons aujourd'hui et vous allez y travailler dans peu de temps sur la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle, dont on sait que ce sont des clefs. le travail, libérer l'embauche. C'est nécessaire à la fois pour les employés, mais aussi pour les entreprises. Équité : il nous faut effectivement, dans nos réformes fiscales, contribuer à concilier un certain nombre de mesures qui confortent l'attractivité.

Nous devons surtout agir dans la stabilité et la persévérance, parce que notre politique économique ne portera ses fruits que si elle va jusqu'au bout, notamment concernant la libération de notre potentiel de croissance. Vous vous inquiétez, monsieur le sénateur, du taux de 1,7

une délégation de parlementaires et de fonctionnaires de la commission des lois de l'Assemblée nationale du Koweït, conduite par son président, M. Mohammed Hussein Al Dallal. Ils sont accompagnés par notre collègue Dany Wattebled, président délégué du groupe d'amitié pour le Koweït. Arrivée lundi, la délégation a rencontré, hier, notre collègue Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, pour échanger sur la question des fausses informations ou. Les députés Les députés se sont également entretenus avec plusieurs membres du groupe d'amitié France-Pays du Golfe. Le Sénat français entretient d'excellentes relations avec l'Assemblée nationale du Koweït. Cette visite contribue à les conforter. Dans ce contexte d'intensification de notre coopération interparlementaire, une délégation du groupe d'amitié a d'ailleurs prévu de se rendre au Koweït à l'automne. Mes chers collègues, en votre nom à tous, permettez-moi de souhaiter à nos homologues de l'Assemblée nationale du Koweït la plus cordiale bienvenue et un fructueux séjour. séjour. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,

en 2017. Vous imaginez bien que ce département a été dans l'incapacité financière et organisationnelle d'accueillir un tel afflux de population. J'ai parlé des Hautes-Alpes, mais nous pourrions évoquer le cas de très nombreux autres départements.

en créant un schéma national d'accueil des demandeurs d'asile, afin de fixer la répartition des places d'hébergement destinées aux demandeurs sur le territoire national. À travers ce schéma national se déclinent des schémas régionaux. En effet, l'objectif est double : d'une part, accueillir et héberger dignement les demandeurs d'asile, conformément aux obligations internationales qui nous incombent ainsi qu'à notre tradition républicaine ; d'autre part, répartir équitablement les demandeurs sur l'ensemble du pays, pour éviter que certains territoires, notamment les métropoles, ne soient confrontés à des difficultés d'accueil. En d'autres termes, ce schéma est aussi un mécanisme de solidarité nationale entre les territoires. Comment ne pas y être favorable quand, parallèlement, une plus grande solidarité est prônée à l'échelle européenne ? Cependant, l'histoire récente nous apprend que les flux migratoires peuvent varier, et ce sur une période très brève. L'avenir prochain nous fait penser que le nombre de déplacés et de réfugiés, en particulier pour des raisons environnementales, va croître de manière exponentielle. Par conséquent, tout système d'accueil efficace doit faire preuve de souplesse et, surtout, être capable de s'adapter aux éventuels changements d'échelle. De fait, adapter le schéma national et les schémas régionaux régionaux qui en résulteront, c'est aussi aider les élus locaux qui gèrent au quotidien les demandeurs d'asile et les différents problèmes que ceux-ci peuvent avoir à affronter, singulièrement avec l'administration. Nous ne pouvons les laisser seuls avec ces structures, car c'est tout simplement dépassé eu égard à l'ampleur d'une situation donnée. Je vous propose donc, mes chers

pour toute la durée de l'étude de leur dossier de demande de statut. Cet article prévoit leur hébergement, ainsi qu'un suivi administratif, avec un accompagnement tout au long de la procédure, un suivi social- accès aux soins, scolarisation des enfants ... -et une aide financière alimentaire.

préalablement à l'étude du projet de loi, de nombreuses associations de défense des droits des femmes nous ont alertés sur la condition des demandeuses d'asile, majeures et mineures, dans les centres. Deux problèmes majeurs ont été soulevés. Premièrement, les femmes représentent plus de 30 % des demandeurs d'asile, mais les centres d'accueil ne disposent pas de 30 % de places pour les femmes. Le second problème relevé est le traitement moral et physique réservé aux femmes dans les centres mixtes. Pour pallier ces difficultés, le présent amendement vise à reconnaître et à prendre en compte la spécificité du genre féminin des demandeuses d'asile et à assurer ainsi leur sécurité au sein des CADA, en prévoyant des places d'hébergement qui leur seraient spécifiques. La parole

Le présent amendement vise à réserver des places d'hébergement spécifiques pour les femmes dans les CADA. Vous savez sans doute que les migrants sont presque tous des personnes vulnérables. Cependant, dans cette vulnérabilité, il est une vulnérabilité spécifique,

ces structures sont mixtes, les conditions nécessaires à ce que ces femmes puissent se reconstruire. C'est la raison pour laquelle l'amendement vise, comme celui qu'a présenté ma collègue voilà un instant, à réserver, dans les CADA, des places spécifiques en non-mixité

préalablement à l'examen du projet de loi qui nous occupe aujourd'hui, nous avons également eu l'occasion de dialoguer avec le milieu associatif

évidemment, tous les exilés sont aujourd'hui dans une situation de précarité déplorable. L'environnement de ceux qui ont fui leur pays d'origine du fait des du fait des persécutions qu'ils y subissaient au titre de leur orientation sexuelle mérite toutefois une attention toute particulière. Il n'est pas acceptable que les personnes LGBTI, que notre commission nomme « personnes homosexuelles », subissent, dans les CADA, des persécutions et violences, tant morales que physiques, similaires à celles auxquelles elles ont été confrontées dans les États qu'elles ont fuis. Le présent amendement tend ainsi à la création, au sein des CADA, de places d'hébergement spécifiques pour les personnes mineures et majeures LGBTI, afin que soit assurée leur sécurité, lorsque celle-ci n'est pas garantie.

Comme vous le savez, les demandeurs d'asile qui ne sont pas hébergés disposent d'un pécule.

entend par « conditions matérielles d'accueil, les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons,

Peut-être le problème sera-t-il moins aigu si nous allons effectivement vers cette déconcentration. est ainsi libellé : La parole est à M. Fabien Gay. Le présent article prévoit que l'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence du demandeur d'asile en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ce faire, le préfet devra tenir compte de la situation personnelle et familiale du demandeur, de son état de vulnérabilité, comme cela a été inséré en commission, de ses besoins et de l'existence de structures permettant sa prise en charge.

Nous estimons que le pouvoir administratif ne doit pas disposer d'une telle prérogative et que le choix de la région de résidence, argumenté et justifié, doit garantir aux demandeurs d'asile la proximité avec leur famille, notamment leurs enfants, ainsi qu'avec les soutiens ainsi qu'avec les soutiens bénévoles qui les accompagnent et les assistent. Il s'agit également de prendre en compte l'état de santé du demandeur en ne l'éloignant pas des structures qui lui procurent des soins. Ces obligations fondamentales doivent être prises en compte, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans le considérant 28 de son avis.

se rendre à un entretien, se présenter aux autorités ou fournir les informations utiles, par exemple -peut répondre à un motif légitime. La suppression de cette mention par le projet de loi supprime la marge la marge d'appréciation de l'OFII, qui ne pourra plus évaluer si une absence à un entretien ou une non-présentation aux autorités se justifie par un motif légitime. L'amendement

est à M. Rachid Temal. Il s'agit d'un amendement de coordination relatif à l'information du demandeur d'asile visant à supprimer la mention du caractère de plein droit du refus ou du retrait des conditions matérielles d'accueil. Nous voulons revenir sur le caractère automatique du refus des conditions matérielles d'accueil.

pouvant justifier que le demandeur n'ait pu se rendre à son entretien ou n'ait pu se présenter aux autorités dans les délais et conditions qui lui avaient été fixés. Alors même qu'il pourrait faire valoir une raison légitime, les conditions matérielles d'accueil lui seront retirées immédiatement et de plein droit. D'autre part, ce caractère automatique du retrait ne permet plus de prendre en compte la vulnérabilité du demandeur. On ne peut avoir à la fois l'automaticité du retrait des conditions matérielles d'accueil et la prise en compte de la vulnérabilité. Le caractère automatique du retrait contredit donc la deuxième phrase de l'alinéa 41 qui vise justement à garantir qu'une « décision de retrait des conditions matérielles d'accueil [ ...] prend en compte la vulnérabilité du demandeur

Cet amendement vise en effet à supprimer la disposition selon laquelle les schémas régionaux d'accueil des demandeurs d'asile définissent les actions à mener pour assurer l'éloignement des déboutés du droit d'asile et les transferts des personnes sous procédure Dublin. les schémas régionaux d'accueil ont aujourd'hui pour objet d'organiser les conditions matérielles d'accueil concernant l'hébergement et n'ont certainement pas vocation à intervenir en matière d'éloignement. Une telle disposition traduirait une grave confusion des genres : ces schémas ne sont pas des outils au service de l'éloignement des déboutés du droit d'asile.

qui soit conforme à un schéma national. Il est soumis, ce qui est tout à fait cohérent, à l'avis- donc, c'est un sujet de concertation -du comité régional du logement. Or le groupe

sur l'adoption d'un schéma régional qui dépend lui-même d'un schéma national. Je m'en remets à votre réflexion. Toutefois, si le comité régional du logement émet un avis conforme négatif, il ne peut y avoir de schéma régional.

ne peut avoir lieu puisque, du coup, on prive l'État de son pouvoir prescriptif. Je ne sais pas si c'est l'intérêt de la région, de ses collectivités et, bien entendu, des personnes qu'il s'agit d'héberger et d'accueillir.

à un vote par scrutin public sur un sujet qui n'a peut-être pas été complètement vu, je suggère de prendre un instant de réflexion. dans le droit fil de l'intervention de notre collègue Alain Richard et de mon explication de vote précédente. Eu égard à l'importance du sujet et qui conduit finalement à importer en France les difficultés européennes en matière de répartition

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande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

9, afin que le décret en Conseil d'État qui devra définir les normes minimales en matière de prestations et d'accompagnement social garantisse la qualité des prestations délivrées et l'adéquation de l'accompagnement aux besoins des demandeurs d'asile.

il est compréhensible que, dans un premier temps, nos préoccupations portent d'abord sur la quantité d'hébergements disponibles. M. le rapporteur l'a rappelé, les solutions d'hébergement sont encore insuffisantes et de nombreux demandeurs d'asile occupent des hébergements d'urgence de droit commun.

Monsieur le ministre

L'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'accueil en lieu d'hébergement des demandeurs d'asile est assuré pendant la période d'instruction de la demande et, le cas échéant, jusqu'au transfert vers un autre État. Il prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'OFPRA ou lors de la notification de la CNDA, soit dans un délai d'un mois, que le Gouvernement, je vous Nous souhaitons, pour notre part, que l'accueil en hébergement des demandeurs d'asile court jusqu'à la fin du deuxième mois suivant l'expiration du délai de recours contre la décision de l'OFPRA ou la notification de la décision de la CNDA. Il s'agit là d'une mesure humaine permettant aux déboutés du droit d'asile de bénéficier d'un accueil digne, afin de demander leur admission au séjour à un autre titre. Cet amendement s'inscrit également en cohérence avec notre volonté de revenir sur l'article 23 du texte, qui prévoit que la démarche pour un autre titre de séjour doit être effectuée en parallèle à la demande d'asile. Nous y sommes opposés, un tel dispositif portant atteinte aux droits de certaines catégories de demandeurs d'asile, notamment les personnes « dublinées

comme seuls refuges de fortune après un voyage souvent épuisant et traumatisant pour les exilés. Il est scandaleux que des familles entières se retrouvent à vivre dans ces conditions. Certains s'en émeuvent en pensant à la dégradation de l'image touristique de notre pays, loin d'eux bien sûr l'idée du respect de la dignité humaine, qui est ici bafouée. Je n'épiloguerai pas sur l'exemple emblématique du campement de la Villette. Il est désormais urgent de s'interroger sur les dispositions à mettre en place pour assurer à ces exilés un accueil digne. Cela passe par des conditions matérielles d'accueil bien encadrées et par l'allocation de moyens, qui leur permettent de subvenir à leurs besoins primaires, en attente de mieux. Or, au même titre que l'hébergement, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile est souvent retardé, faute de moyens administratifs suffisants. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que la situation des demandeurs d'asile concernés se dégrade. C'est d'autant plus problématique que l'interdiction de salariat court sur une période de neuf mois. C'est pourquoi nous proposons au travers de cet amendement de prévoir un délai de huit jours maximum pour que le versement de l'allocation pour demandeur d'asile soit effectué. Il est urgent de répondre aux dysfonctionnements actuels en matière de retards et de délais. En outre, nous souhaitons supprimer l'arrêt du versement de l'ADA un mois après l'audience publique de la CNDA. Comme le Conseil d'État l'a noté, ce délai est beaucoup trop court pour permettre aux personnes concernées et aux associations qui les accompagnent dans leurs démarches d'organiser leur départ des lieux d'hébergement

le versement de l'ADA serait supprimé au terme du mois au cours duquel la décision de la CNDA a été lue en séance et non plus notifiée. Ces trois amendements visent à allonger ce délai,

Il est totalement illusoire d'imaginer qu'il sera plus facile d'éloigner une personne qui vient d'être déboutée, alors même qu'on ne saura pas où elle est. Il est donc assez logique de proposer

La commission a donc conditionné le maintien dans les lieux d'hébergement à une décision motivée de l'autorité administrative. Ce dispositif a d'ailleurs déjà été adopté au Sénat en 2016. J'insiste sur ce point, le débouté pourra rester temporairement dans son lieu d'hébergement pour trouver une solution alternative. Toutefois, la procédure sera beaucoup mieux encadrée.

? Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements. En effet, il ne nous semble pas possible de faire en sorte que la personne déboutée

Le scrutin est ouvert.

de quitter son lieu d'hébergement. L'affaire est alors portée devant le tribunal administratif, qui statue en référé. Cette procédure reste peu utilisée, alors même que les dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile sont engorgés et que des déboutés s'y maintiennent indûment. indûment. Cet amendement vise donc à permettre au gestionnaire du centre d'hébergement de saisir lui-même la justice lorsqu'un débouté du droit d'asile refuse indûment de quitter les lieux et à prévoir une compétence liée du préfet et du gestionnaire pour s'assurer de la mise en oeuvre de cette procédure.

Avec cette circulaire, l'État a déjà recensé 4 000 personnes dans les centres et hôtels sociaux, en y envoyant des « équipes mobiles », constituées d'agents des préfectures et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le Gouvernement se justifie en estimant qu'il s'agit d'un moyen indispensable pour orienter les publics en fonction de leur situation - réfugiés, déboutés ou autres - et désengorger des centres saturés. Pour notre part, nous ne pouvons pas ne pas nous inquiéter du sort des personnes en situation irrégulière qui ont le droit, sous une forme ou une autre, de bénéficier d'un hébergement. Nous estimons ainsi que ces mesures contreviennent au principe de l'inconditionnalité de l'accueil prévu par le code de l'action sociale et des familles, mais aussi par la loi DALO, aux termes de laquelle les personnes en situation irrégulière, sans pouvoir prétendre à un droit au logement, peuvent être désignées par les commissions de médiation aux fins d'obtenir un hébergement. Au-delà du droit, c'est un principe d'humanité qui est en cause. Alors que de nombreux citoyens et citoyennes se mobilisent partout, en France, individuellement ou dans le cadre des associations, pour venir en aide à ces personnes qui ont fui la guerre et la misère au péril de leur vie, on attend de l'État qu'il accompagne la solidarité et non qu'il vienne l'entraver. La parole est à M. Rémi Féraud,

un problème de principe lié à l'inconditionnalité de l'accueil et au fait que les associations ou les structures qui gèrent l'hébergement d'urgence ne doivent pas sortir de leur rôle

Même avis défavorable. Comme le Président de la République et le Premier ministre ont eu l'occasion de le dire, si l'accueil doit être inconditionnel, il ne doit pas être indifférencié.

à supprimer un cas supplémentaire de retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans le cas où le demandeur aurait présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, en raison des effets pervers que cette disposition pourrait engendrer.

de sa situation ou lorsqu'elle présente sa demande d'asile au-delà du délai légal de 120 jours. Il nous semble que cet alinéa soulève des difficultés. D'abord, il est quand même étrange de priver de droit un étranger alors même qu'il a le droit de demander le réexamen de son statut : il y a une contradiction dans cette situation. Ensuite, concernant l'expiration du délai-

que le versement de l'ADA peut intervenir près de deux mois après l'accès du demandeur à la plateforme d'accueil. Pour cette raison, nous souhaitons encadrer ce versement par l'instauration d'un délai beaucoup plus court, de huit jours à compter de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil.

explication de vote. Si l'on souhaite accélérer les procédures de demande d'asile, il est absolument indispensable que les demandeurs d'asile disposent des moyens qui leur permettent de vivre au moment où

par la mairie de Paris, à la porte de la Chapelle notamment. Les centres de premier accueil offrent un hébergement aux étrangers en situation irrégulière, quelle que soit cette situation. Des services d'accompagnement juridique seront mis en place afin de faciliter le dépôt d'une demande d'asile pour ceux qui en ont exprimé la volonté. Il s'agit

a cessé d'assurer cette orientation d'aval, et dès lors que le centre a fermé, les campements de rue se sont reconstitués. Permettre aux communes de mener cette action, leur donner la légitimité de la loi,

aux petits éléments donnés par le rapporteur, qui a dit qu'il existe déjà des CAES. Non ! On voit bien qu'ils ne remplissent pas cette fonction.

Beaucoup de communes le demandent ; elles veulent prendre des responsabilités. Que la loi leur donne cette possibilité

Vous savez bien que 70 % des demandeurs d'asile seront déboutés du droit d'asile, si bien que nous avons à traiter un problème massif, qui est un problème de société : c'est que le demandeur d'asile n'a généralement pas droit à l'asile. Nous allons naturellement lui permettre de défendre ses chances, et nous faisons en sorte que des garanties lui soient apportées. Mais nous ne pouvons pas nous mettre systématiquement du côté du demandeur d'asile, comme si sa demande allait être probablement admise, alors que nous savons que la réalité est que, dans 70 % des cas, elle ne le sera pas. Le problème que nous avons à traiter ici, qui est le problème principal, n'est pas de construire un système de garanties supplémentaires pour les demandeurs d'asile, ... Non ! C'est un problème de protecteur qui remplit intégralement nos obligations internationales. Le problème d'aujourd'hui, la question qui nous est posée, que la réalité nous impose de traiter, est celle de

besoin pour traiter les demandes d'asile légitimes ! Vous n'avez pas lu l'amendement ! Ce débat sous-jacent, il faut quand même réussir à le formuler ; sinon, vous allez continuer à vous faire les porte-étendards du demandeur d'asile qui sera débouté, tandis que nous allons continuer, sans le dire- mais nous devons aussi l'assumer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

des règles de délivrance de la nationalité française. Nous devons pouvoir choisir au cas par cas qui aura la chance, pour ne pas dire l'honneur, de devenir Français. Cet amendement vise à supprimer tous les articles de notre législation qui consacrent le droit du sol. Je le rappelle pour mémoire, l'un de nos anciens collègues, alors ministre de l'outre-mer, avait déclaré

de modifier le code de la nationalité. Cette proposition a bien sûr été refusée par le Président de la République de l'époque, grand architecte de l'immigration de masse, M. Chirac, avant d'être frappée d'inconstitutionnalité. On ne peut évidemment pas avoir un droit du sol en métropole et un droit du sang dans nos collectivités d'outre-mer. Mes collègues à l'Assemblée nationale ont déposé une proposition de loi constitutionnelle qui est au fondement de notre contre-projet. Nous souhaitons inscrire dans la Constitution une mesure que nous considérons comme préalable à toute politique d'immigration.

Le code civil distingue l'attribution et l'acquisition de la nationalité française. L'attribution de la nationalité française vise ceux qui naissent français.

Le code civil distingue en outre plusieurs modes d'acquisition de la nationalité française visant ceux qui, ayant une nationalité étrangère, deviennent ensuite français. Il prévoit notamment l'acquisition par la naissance et la résidence en France, la nationalité étant acquise à la majorité de l'enfant. Elle peut faire l'objet d'une déclaration anticipée de la part du mineur de plus de seize ans, ou formée par les parents au nom de l'enfant à partir de ses treize ans.

fiches S. Subordonner le droit de la nationalité aux fiches S est proprement insensé, pour une raison que nous devons constamment rappeler : l'immense majorité des personnes qui sont fichées S n'ont commis aucune infraction, aucun délit, aucun crime. C'est un fichier qui qui fait partie des outils du renseignement, outils utiles, car le renseignement est nécessaire dans la lutte contre le terrorisme. Cela procède d'un certain nombre de déclarations politiques

là, me semble-t-il, les dangers d'un texte sur l'immigration, l'asile et l'intégration dans lequel on voudrait insérer des amendements

L'enfant né en France de parents étrangers n'acquiert pas d'office la nationalité française. Il l'acquiert à la majorité,

de bien le comprendre : ce qui définit la communauté nationale, ce sont les dispositions du code civil relatives au droit de la nationalité. Notre conception du droit du sol

telle instrumentalisation de ce département, qui connaît des difficultés majeures, pour faire passer des idées abjectes et nauséabondes m'indigne profondément Cet amendement n'a rien à voir avec ceux que je défendrai tout à l'heure et qui s'expliquent par une situation bien particulière, partagée sur aucun autre territoire.

condition de résidence pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans ; possibilité de décliner la qualité de français dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent de réclamer à partir de seize ans la nationalité française par déclaration s'il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans ... Et la liste des cas, des exceptions et des conditions n'est pas exhaustive

jusqu'où va l'imagination débordante de certains d'entre vous pour compliquer la vie d'enfants parfaitement intégrés sur notre territoire, pour les stigmatiser en les renvoyant aux conditions de vie de leurs parents dix-huit ans plus tôt ! C'est vraiment invraisemblable ! Pour notre part, nous pensons que toutes ces conditions d'accès à la nationalité française pour l'enfant mineur né en France de parents étrangers sont inappropriées, en contradiction avec l'intérêt supérieur de l'enfant et, surtout, contraire à nos valeurs républicaines. La France n'est pas une réalité ethnique. C'est l'existence d'un destin commun qui doit fonder l'accès à la nationalité.

! Quoi qu'il arrive- je crois que le sujet le mérite -, la flamme de la Résistance française ne doit pas s'éteindre, et ne s'éteindra pas ! Charles Pasqua était de cette espèce d'hommes d'État guidés par le bien commun et par l'intérêt supérieur de la Nation. Charles Pasqua savait précisément ce que voulait dire être ou devenir français. L'amendement que nous vous proposons s'inspire directement d'une loi qu'il a défendue ici, en 1993. Aujourd'hui, l'article 21-7 du code civil prévoit qu'un enfant né de parents étrangers acquiert automatiquement la nationalité française à sa majorité

de préciser que le jeune étranger souhaitant devenir français doit avoir manifesté sa volonté d'intégrer la communauté nationale par une démarche individuelle et active. Mes chers collègues, ce principe est d'une importance capitale. Nous devons affirmer que la nationalité n'est pas une pochette-surprise que l'on reçoit à sa majorité ! La nationalité se mérite, mais elle doit aussi se vouloir. Voilà ce que nous vous proposons de voter ! Est français qui reconnaît que la loi de la République est la seule qui s'applique sur le territoire de la Nation

rectifié et 31 rectifié sont issus d'une proposition de loi que j'ai déposée le 25 avril dernier et sur laquelle j'ai souhaité que le Conseil d'État rende un avis, compte tenu de la sensibilité du sujet. Le récent soulèvement populaire qui a eu lieu à Mayotte a relancé la prolifération de prises de position autour de la question du droit du sol dans ce département et, plus généralement, de sa remise en cause dans notre pays. Il existe à Mayotte des raisons objectives et insoutenables qui ne se retrouvent sur aucune autre partie du territoire français et qui justifient aujourd'hui ce débat et le dépôt de tels amendements. Sur une compréhension illusoire de la manière dont on acquiert la nationalité française, des femmes, majoritairement de nationalité comorienne, viennent à Mayotte dans des conditions de voyage précaires et dangereuses, afin d'y accoucher. En 2007, 10 000 nouveau-nés ont vu le jour au centre hospitalier de Mayotte, et 74 % de ces enfants sont nés de mère étrangère et la moitié de deux parents étrangers. Cette chimère d'un droit du sol automatique pousse encore un nombre considérable de parents à laisser leur enfant à Mayotte lorsqu'ils font l'objet d'une mesure d'éloignement.

telle pression migratoire insensée entraîne des conséquences en matière d'ordre public. Elle a des effets sur tous les services publics, notamment la santé et l'éducation nationale. Voilà la réalité de notre situation sur place ! Est-il digne de notre République de laisser cette situation perdurer ? Je ne le pense pas. C'est la raison pour laquelle je présente ces deux amendements. L'amendement n° 30 rectifié exige que l'un des parents d'un enfant né à Mayotte ait été présent de manière régulière sur le territoire national depuis plus de trois mois

si l'un des parents au moins la remplit effectivement. Ces amendements n'apportent aucune dérogation limitée aux modalités d'acquisition de la nationalité française. Ils ne remettent pas en cause le principe de la naturalisation par l'effet de la résidence en France et ne modifient pas la durée de résidence exigée. Ils maintiennent également la possibilité pour un enfant né de parents étrangers de résider sur l'ensemble du territoire national, à Mayotte comme sur le reste du territoire, cette résidence comptant pour le bénéfice de la naturalisation. Le contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité auquel le Conseil d'État les a soumis devrait, je l'espère, vous convaincre de leur légitimité. J'en conviens, leur adoption ne viendra pas seule à bout de la difficulté. Mais elle permettra une respiration. je compte sur vous pour voter en faveur de ces amendements. Je compte également sur la population pour adopter localement des comportements responsables qui viendront à bout des pratiques frauduleuses.

tel amendement me semble contraire à notre tradition juridique, en vertu de laquelle la naissance en France n'est pas à elle seule attributive de nationalité- nous venons de l'évoquer -, mais doit être confortée par d'autres éléments de rattachement. La commission émet donc un avis

jugée parfaitement conforme à la Constitution. Je rappelle à notre assemblée qu'il s'agit d'une adaptation limitée de l'un des aspects du droit du sol, dans un contexte de pression migratoire sans précédent. Il est prévu d'exiger, pour l'acquisition de la nationalité des enfants nés à Mayotte de parents étrangers, que l'un des parents ait été présent de manière régulière sur le territoire national depuis plus de trois mois

Comme l'a relevé le Conseil d'État en s'appuyant sur les données de l'INSEE, 41 % des résidents à Mayotte sont de nationalité étrangère, dont la moitié en situation irrégulière. Le taux de natalité est de 40 pour 1000, contre 12 pour 1000 pour le territoire métropolitain. En 2016, 74 % des enfants sont 74 % des enfants sont nés de mère étrangère, le plus souvent comorienne. Le Conseil d'État considère que ces éléments constituent des caractéristiques et des contraintes particulières. L'amendement répond donc parfaitement aux dispositions et au cadre fixé par l'article 73 de la Constitution, qui permet d'adapter les lois aux caractéristiques et contraintes particulières des départements ultramarins.

mélangé les deux questions, nous aurions vu fleurir une série d'amendements qui, de proche en proche, auraient pu remettre en cause ce qu'est aujourd'hui le droit de la nationalité.

que cette proposition s'inscrit dans une série d'actions que mène aujourd'hui le Gouvernement vis-à-vis des autorités comoriennes. Comme vous le savez, il existe une pression extrêmement forte de la part de la diplomatie française sur l'État comorien pour qu'il respecte un certain nombre de règles. En outre, les difficultés de Mayotte ne se limitent pas au seul problème de la nationalité, mais concernent toute une série d'infrastructures sur lesquelles le Gouvernement a fait des propositions d'ensemble. Si Thani Mohamed

et la nation française, je disais simplement que l'État français a eu une conception de la nation française qui n'est pas la nôtre. Je rappelle que l'État français- Vichy -a déchu de leur nationalité 15 000 Français juifs Il a ensuite décidé de ne pas accorder la nationalité française aux enfants juifs nés en France de parents étrangers. C'est à ce titre que je soutiens une autre idée de la citoyenneté française. La

de la nationalité. Je respecte beaucoup le travail qui a été fait par M. le vice-président Mohamed Soilihi sur son territoire pour essayer de trouver une solution. Je sais le temps qu'il y a consacré, la réflexion qu'il a menée, la prudence avec laquelle il aborde ce sujet.

Conseil d'État, je le rappelle, n'est pas le Conseil constitutionnel. Il justifie la possibilité de cette dérogation pour le territoire sur le fondement l'article 73 de la Constitution, en raison des caractéristiques du territoire. Rien ne dit que le Conseil constitutionnel aurait le même avis. également dans son avis que « eu égard à l'objet de la proposition de loi, le Conseil d'État relève plus généralement l'intérêt que soit menée une campagne d'information à Mayotte et aussi à destination des pays d'origine des personnes y immigrant irrégulièrement sur l'état du droit qui résulterait du vote de la proposition de loi ». Cela signifie que votre proposition de loi, cher collègue,

aussi. Les dispositions spécifiques et restrictives de circulation des étrangers à Mayotte par rapport à l'Hexagone renforcent encore la difficulté de la situation.

Je pense sincèrement qu'il se trompe, car ils ouvrent une brèche pour toutes celles et tous ceux qui veulent remettre en cause le droit du sol. Ce sont des amendements qui enfreignent le principe fondamental de l'intérêt de l'enfant. Ils ouvrent aussi une brèche dans l'unicité de notre Je connais Mayotte pour m'y être rendue il y a quelque temps, et je sais que les Mahoraises et les Mahorais vivent une situation très difficile, que personne ne doit ignorer. Toutefois, je ne pense pas

Nous suivons, bien sûr, les éléments d'actualité. Je ne vous cache pas, cher collègue, que nous avons tous été impressionnés par vos explications, par leur caractère, semble-t-il, adapté aux problèmes rencontrés à

d'inscrire votre proposition de loi, cher collègue, à l'ordre du jour, dont le Gouvernement a la maîtrise, à la fois au Sénat

d'ici. C'est ouvrir une brèche que de faire une République qui n'est plus universelle, mais qui est à plusieurs vitesses. La France, la République, doit rester ce qu'elle est.

la Nation que nous sommes, qui fait l'honneur de la France. Monsieur le ministre d'État, je ne partage pas souvent vos idées, vous ne l'ignorez

La départementalisation qui a été voulue par le gouvernement de l'époque, en 2011, est un échec. Vous l'avez votée ! C'est un échec parce que la République n'a pas été à la hauteur des besoins de ce territoire. Je tiens à le dire, si aujourd'hui la plus grande maternité française est Mamoudzou, c'est parce que des femmes, notamment de la Grande Comore, estiment que, quoi qu'il arrive, il vaut peut-être mieux venir accoucher sur le territoire national.

dramatique, la solution qu'il propose n'est pas une bonne réponse. Nous souhaitons naturellement que le droit de la nationalité ne soit pas touché par les

ce texte. Si ces amendements étaient adoptés, que pourrions-nous dire à propos d'amendements identiques sur la Guyane, en lien avec le Surinam ?

l'accent sur une situation dramatique, qui fut rappelée en son temps par notre ancien collègue M. Baroin, qui, encore une fois, s'était

parler de « génocide par substitution »- ce n'est pas moi qui l'ai dit le premier ! Quand on réussit à se libérer de ses dogmes, quand on réussit à voir la réalité en face, quand on habite la planète Terre, eh bien on fait comme les Mahorais

cette proposition sur Mayotte, c'est évidemment parler de la Guyane et remettre en cause l'acquisition de la nationalité. Évidemment

Le problème, c'est que tous les jours des bateaux appelés kwassa-kwassa transportent des gens, au péril de leur vie, pour arriver de manière illégale. Il s'agit de passeurs qui oeuvrent dans l'illégalité la plus complète grâce à des connivences et à de la corruption. Il faut l'empêcher, ce qui ne pourra se faire que si la République française passe un accord avec les Comores : il n'y a pas d'autre solution,

a lancé cette semaine un groupe de réflexion sur l'immigration clandestine. C'est très bien, mais l'heure n'est plus tellement aux groupes de réflexion,

L'article 73 de la Constitution permet qu'une législation différente s'applique suivant les territoires ultramarins. Je fais observer à certains collègues que, depuis vingt ans, sous un gouvernement auquel j'avais l'honneur d'appartenir, il a été décidé que le droit du suffrage serait différent en Nouvelle-Calédonie de ce qu'il est dans le reste du pays : c'est en vigueur et c'est constitutionnel ! Donc, il y a un motif d'intérêt général, que le Conseil d'État a parfaitement résumé, pour empêcher l'acquisition de la nationalité française dans des conditions désordonnées sur ce territoire. Je veux aussi souligner que l'idée,

Le problème ne fait que s'aggraver à Mayotte. Nous avons une opportunité et nous avons, constitutionnellement un lien avec l'objet du texte, pour amender maintenant dans ce sens. C'est licite, légitime, nécessaire et équitable

d'une minorité qui se sert de nos territoires comme d'un fonds de commerce. C'est inacceptable ! Je me demande même s'ils savent où se trouvent la Guyane et Mayotte, parce qu'ils sont souvent fâchés avec la géographie

Soilihi prend ses responsabilités et nous respectons ses amendements. Nous ne les avons pas signés, parce que nous ne sommes pas dans la même situation. Nous sommes une nation arc-en-ciel. Je suis, quant à moi, le pur produit de cette nation arc-en-ciel.

J'ai écouté vos propos et je suis, à titre personnel, tenté de vous suivre. Mais j'ai le plus profond respect pour le travail qui se fait ici, au Sénat.

a bien voulu s'en remettre à la commission des lois : c'est la réponse qu'il apporte à la demande de M. le ministre d'État de retrait de son amendement.

ce qui lève toute ambiguïté et tout embarras pour son auteur. Par conséquent, notre assemblée peut, en tout état de cause, se prononcer sereinement sur ce problème, sans que notre collègue ait à en assumer seul la responsabilité. Il me semble important que nous réglions dès à présent cette difficulté. J'ai beaucoup apprécié la la réponse très mesurée que M. le ministre d'État nous a faite. J'interprète cette réponse comme un encouragement à faire aboutir cette réforme pour Mayotte : il pour Mayotte : il ne se serait pas engagé à ce que, en cas d'échec du processus sur ce point dans le cadre de la loi sur l'immigration, le Gouvernement inscrive à son ordre du jour prioritaire

explication de vote. Le plus souvent, je trouve que les explications de vote ne sont pas forcément nécessaires, mais, en l'occurrence, la situation est très particulière. Je connais bien la situation de la protection de l'enfance à Mayotte. Elle est indigne de la République,

vous le savez, ma part de responsabilité et de culpabilité dans cette affaire. Pour autant, je comprends aussi l'appel au secours

faites un projet de loi ! Que le Gouvernement prenne ses responsabilités à l'issue de ce débat pour apporter aux élus de Mayotte, à sa population et aux enfants la protection et la dignité auxquelles ils ont droit ! Je mets aux

Le scrutin est ouvert.

Nous l'avons déjà affirmé, notre objectif est de réduire drastiquement les flux migratoires afin d'aboutir à un solde annuel de 10 000 entrées. Pour y parvenir, il est nécessaire de contrôler beaucoup plus strictement la délivrance des visas, lesquels permettent à certains étrangers entrés légalement de se maintenir clandestinement sur notre territoire une fois la validité du visa expirée. En effet, sur près de 135 000 personnes régularisées, quelque 68 000 seraient entrées un visa de tourisme. Alors oui, il est essentiel d'encadrer de façon beaucoup plus restrictive l'octroi des visas. C'est tout l'objet du présent amendement, qui prévoit la possibilité de subordonner leur délivrance au paiement d'une taxe, ainsi qu'au dépôt d'une caution couvrant les frais de rapatriement, caution restituée par l'autorité consulaire au retour de la personne sollicitant le visa dans l'état d'origine. Ce dispositif ne serait évidemment pas automatique, mais applicable selon les États en vertu d'une liste établie annuellement par décret, après avis des commissions parlementaires compétentes et organisation d'une procédure de consultation publique.

sous la mandature de Nicolas Sarkozy, il est entré plus d'étrangers en France que sous le gouvernement Jospin. Une prouesse qui mérite d'être rappelée ! Cela rend de plus en plus permissives les conditions du droit au séjour, qui ne tiennent compte ni des capacités d'accueil de notre pays ni des nécessités de son économie. Vous savez très bien qu'un titre de séjour n'est, par définition, qu'une autorisation temporaire de demeurer sur le territoire national, une autorisation donnée par les Français à des étrangers. Un étranger présent sur le sol français sans titre de séjour est en situation irrégulière. Il doit, s'il n'est pas éligible au droit d'asile, être reconduit dans son pays d'origine. Le système actuel- votre système ! -favorise la fraude et pèse sur les finances publiques puisque les rapatriements sont à la charge de l'État, c'est-à-dire de nos compatriotes. Nous proposons à travers cet amendement de subordonner l'obtention d'un titre de séjour au paiement d'une taxe, ainsi qu'au dépôt d'une caution visant à couvrir les frais de rapatriement. Il s'agit, là encore, d'une mesure de bon sens : il ne faut pas que l'éventuel rapatriement de ces étrangers soit uniquement financé

mais je souhaite apporter un premier éclairage sur les conséquences d'une telle remise en cause. Toutes les associations membres de l'Observatoire du droit à la santé des étrangers, l'ODSE, sont unanimes : le respect des droits réservés aux étrangères et étrangers malades, droits notamment encadrés par la loi du 11 mai 1998 introduisant la régularisation pour raisons médicales, est mis à mal

Ce dernier étant davantage animé par des objectifs de contrôle des flux que par la préservation de la santé publique, nous nous étions fermement opposés à cette mesure absolument révélatrice de la logique comptable, déjà portée par le gouvernement précédent, en matière de politique migratoire. Nos collègues socialistes ont regretté, dans leur motion tendant à opposer la question préalable, que les mesures de cette loi de 2016 n'aient pas encore pu produire leurs effets. Pourtant, sachez que les premiers chiffres disponibles sont éloquents : le nombre de titres de séjour délivrés pour soins a chuté de 37 % entre 2016 et 2017. Le texte de 2016 a donc ouvert la brèche, et le gouvernement En Marche s'y engouffre. Ainsi, par exemple, l'article 20 du texte que nous examinons prévoit qu'un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement fondée sur le rejet de sa demande d'asile ne pourrait plus solliciter un titre de séjour hors du délai fixé, sauf « circonstances nouvelles ». Cela vise de nombreux étrangers malades, car une part importante des déboutés du droit d'asile relèvent de la procédure du droit au séjour pour soins, comme le révèle le rapport sur l'admission au séjour des étrangers malades.

C'est une mesure que je considère comme injuste, presque cynique, d'une certaine manière. Monsieur Karoutchi, je vous rappelle que, entre 2010 et 2011, pas moins de trois lois avaient modifié le dispositif de l'aide

Il avait également soumis la prise en charge des frais hospitaliers lourds, au-delà de 15 000 euros, à une autorisation préalable de la caisse primaire d'assurance maladie.

Ce renchérissement a conduit des personnes en grande difficulté à renoncer à se faire soigner, ou à reporter leurs demandes de soins.

Pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge, les étrangers en situation irrégulière doivent résider sur notre territoire « de manière ininterrompue depuis plus de trois ans », et leurs ressources ne doivent pas dépasser un certain seuil.

nous en sommes donc à débattre d'une mesure qui figurait en bonne place dans les programmes de François Fillon et de Marine Le Pen Nous le savons, lors du conseil interministériel consacré à l'intégration des étrangers, qui s'est tenu le 5 juin dernier, M. Gérald Darmanin s'est montré favorable à la suppression de l'aide médicale de l'État,

aux problèmes sociaux, aux difficultés administratives, et qui sont souvent dans un état de santé déplorable. La santé est un bien universel et commun. Les ressortissants étrangers doivent pouvoir bénéficier, au même titre que les ressortissants français, de notre système de protection de la santé. Nous ne devons rien céder sur ce point

doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. » La réforme proposée placerait donc les médecins et les personnels soignants face à une injonction paradoxale,

Pour mémoire, l'AME est une aide fournie aux étrangers présents en France, en situation irrégulière, depuis plus de trois mois. Depuis plusieurs années, le nombre de ses bénéficiaires connaît une hausse sensible.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est ouvert.